titulaires à des points de bonification pour l'obtention des diplômes de l'enseignement secondaire- Dès l'âge de 16 ans, en effet, les jeunes peuvent obtenir divers certificats dans le domaine sportif. À titre d'exemple, je citerai le certificat d'initiative fédérale en canoë-kayak, le certificat fédéral de football 1, le brevet fédéral « découverte-initiation » en rugby. Démocratiser le sport en France, c'est en encourager la pratique, mais c'est aussi encourager l'engagement des jeunes au sein de leur propre club, engagement qui mériterait

de pratique. Il est notamment proposé de dégager un temps spécifique au sein de la formation, pour répondre aux enjeux particuliers du sport. Par ailleurs, les sportifs de haut niveau contribuent au rayonnement international de la France et à son attractivité

étudiantes. Concernant le financement des projets développés par ou pour des établissements d'enseignement supérieur, on pourrait tendre vers une organisation territoriale des capacités de sport et favoriser les projets finançables par la contribution vie

En effet, si les enseignants d'EPS, actuels et futurs, sont des dépositaires de l'activité sportive, ils ne sont pas à proprement parler des acteurs participant à la structuration de la politique sportive à l'échelle des territoires comme peuvent l'être l'État, les collectivités territoriales, les fédérations sportives ou certains acteurs économiques.

Rappelons que la nouvelle gouvernance territoriale du sport doit promouvoir une démarche partenariale, afin notamment de mieux identifier les carences dans l'offre locale d'activités physiques et sportives, ainsi que les lieux manquant d'équipements et de sites. Le développement de l'usage du vélo comme moyen de transport est bénéfique en matière de lutte contre les sédentarités et profite à la santé. Il peut aussi offrir, dans certains territoires, une alternative au manque d'équipements strictement dédiés au sport. Aussi, il convient de mentionner dans le périmètre des projets sportifs territoriaux la nécessité de développer des parcours sécurisés de cycles et de marche. mention de cet objectif exprimerait de façon transversale l'ambition inscrite à l'article 1 de la loi du 24 décembre 2019 d'orientation des mobilités, qui recommande notamment « les mobilités actives au bénéfice de l'environnement, de la santé, de la sécurité et de la compétitivité ».

? Comme l'a rappelé M. le rapporteur, le cadre normatif donne déjà compétence aux conférences régionales du sport en matière de lutte contre les violences dans le sport. Ce sujet est effectivement essentiel et ces conférences sont le meilleur lieu pour faire prendre conscience à toutes les parties prenantes de l'importance de ce combat, qui doit nous concerner tous aujourd'hui.

Afin de compléter utilement ces missions, il serait bienvenu qu'elles comportent également un volet environnemental renforcé. Dans sa rédaction actuelle, l'article 4 ne satisfait que partiellement cet impératif, en mentionnant la notion de

s'agit d'exonérer de responsabilités les gestionnaires de sites naturels où se déroulent les activités sportives, uniquement en cas de réalisation d'un risque normal et raisonnablement prévisible. L'article 4 A crée l'article L.

essentiel de ne pas restreindre considérablement les possibilités pour une victime d'agir en responsabilité dès lors qu'un accident serait survenu à l'occasion d'un sport de nature ou d'une activité de loisirs.

Cette précision permet de maintenir l'allégement de la responsabilité des gestionnaires des sites naturels que, comme nous, vous souhaitez, tout en responsabilisant les usagers qui auraient des pratiques dangereuses ou qui exerceraient leur activité sportive dans des espaces naturels non aménagés, en conservant le droit des victimes à obtenir réparation dans certaines situations. Quel est l'avis de la

Par ailleurs, dans sa rédaction actuelle, l'article supprime malencontreusement non seulement la question du renouvellement de la licence pour les majeurs, mais aussi la distinction dans le traitement des mineurs. Or, je vous le rappelle, ceux-ci sont exonérés de la présentation d'un certificat médical en raison des différents contrôles médicaux auxquels ils ont accès aux différents âges de l'enfance, sous réserve bien entendu d'avoir apporté des réponses négatives au questionnaire de santé qu'ils doivent présenter. Dans la démarche de responsabilisation des fédérations voulue notamment dans le cadre de la nouvelle gouvernance du sport, il nous apparaît que les fédérations sont à même de juger des conditions d'exercice des disciplines pour lesquelles elles possèdent la délégation, après avis d'une commission réunissant les personnalités qualifiées. Cet amendement tend d'ailleurs aussi à renforcer la composition de ces commissions médicales.

pour les manifestations sportives transfrontalières. En droit français, les règles applicables pour organiser un événement sportif sont codifiées dans le code du sport : actuellement, pour participer à une manifestation sportive, à défaut de présentation de cette licence, l'inscription est subordonnée à la présentation d'un certificat médical datant de moins d'un an, établissant l'absence de contre-indication à la pratique du sport ou de la discipline concernée en compétition, L'obligation de demander un certificat médical à des participants de pays voisins est peu opérationnelle dans la mesure où ce document est spécifique à la France. Il s'agit donc d'un obstacle important à l'organisation

Si j'entends cet argument sécuritaire, je tiens à souligner que le décret dressant la liste des sports à contraintes particulières n'est pas satisfaisant. C'est pourquoi j'ai proposé à la commission un amendement qui sera examiné dans quelques minutes, afin que ce décret soit pris

pour l'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024, une politique ambitieuse du sport doit être envisagée. Cet amendement vise à compléter l'organisation existante, en intégrant le sport dans le champ des compétences obligatoires des conférences territoriales de l'action publique

Actuellement, cette déclaration comprend des informations relatives aux conséquences sur le changement climatique de l'activité de la société et de l'usage des biens et services qu'elle produit, à ses engagements sociétaux en faveur du développement durable, de l'économie circulaire, de la lutte contre le gaspillage alimentaire, etc. En

présidée alors par Michel Magras. Si l'articulation du parcours sportif avec le parcours scolaire est une nécessité, le « double parcours » étant au coeur de l'accompagnement des sportifs, peu de voies sont ouvertes aux jeunes talents sportifs en échec scolaire, particulièrement en outre-mer. Aussi, nous demandons que soit engagée une réflexion sur la création de parcours « deuxième chance par le sport », afin de ne pas gâcher des potentiels existants et d'offrir à de jeunes sportifs talentueux les opportunités d'encadrement qu'ils méritent.

d'un rapport sur les voies d'accès aux parcours sportifs de haut niveau en outre-mer, avec pour objectif d'éviter le déracinement précoce des jeunes talents. L'Institut national du sport, de l'expertise et de la performance (Insep) étant l'acteur majeur de structuration de la performance et du haut niveau à l'échelon national, c'est à lui que revient ce rôle d'attraction.

aux structures territoriales, et de donner aux structures locales les moyens de s'intégrer à la dynamique et au projet du grand Insep. Vous comprenez ainsi aisément les enjeux : priorité est donnée à la structuration des voies d'accès au parcours sportif de haut niveau en outre-mer, laquelle éviterait le déracinement précoce de nos jeunes talents.

avons structuré les réseaux ultramarins de performance autour de deux établissements publics : un Creps à Pointe-à-Pitre, pour le secteur Antilles-Guyane, et le Creps de la Réunion pour le secteur océan Indien. Ces établissements ont bénéficié d'un renforcement de six postes dans le cadre du déploiement des maisons régionales de la performance, et du transfert des compétences « sport de haut niveau » des délégations En 2022, quatre postes supplémentaires sont fléchés vers l'outre-mer : trois pour la Martinique, un en Guyane. L'objectif prioritaire est de mieux accompagner le parcours des sportifs, depuis la détection jusqu'à l'accès à la

Bien sûr, nous devons tenir compte de ces débats et de leurs conclusions pour leur donner, si possible, une traduction législative, pour ne pas dire un débouché politique.

l'article. Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, cet article est vraiment au coeur du processus de démocratisation du sport, dans la mesure où il s'agit d'accroître la parité au sein des instances nationales et régionales des fédérations. n'est pas seulement symbolique, bien évidemment : il doit être le reflet d'une ambition collective que nous devons porter pour renforcer la place des femmes dans le mouvement sportif et, par là même, impulser une dynamique positive en faveur de la pratique sportive féminine. ce sont 38,8 % des licences sportives qui étaient détenues par des femmes, un pourcentage quasiment identique à la part d'athlètes féminines de haut niveau, qui est de 39 %. En affinant l'analyse, nous pouvons constater que les femmes sont majoritaires dans neuf fédérations seulement, tandis que les fédérations multisports sont beaucoup plus féminisées. En termes de représentativité au niveau des instances des fédérations, des progrès ont été réalisés en faveur de la parité, singulièrement depuis la loi du 4 août 2014 pour l'égalité réelle entre les femmes et les hommes. Le taux de féminisation des conseils d'administration des fédérations olympiques est passé de 27,4 % en 2009 à 42,13 % en 2021. Pour autant, cette évolution n'est pas suffisante et doit être confortée. Le débat que nous allons avoir ne porte pas tant sur le constat, que nous partageons tous, qu'il est nécessaire de tendre vers la parité, mais plutôt sur le rythme à suivre. Pour le dire simplement, nous sommes favorables à une accélération du renouvellement des instances, à la fois nationales et régionales, et des fédérations, dans le sens d'une vraie féminisation.

L'incitation n'a qu'un impact marginal et les dates butoirs placées à des échéances lointaines ne favorisent aucunement le déclenchement d'une dynamique. Nous devons donc nous montrer très proactifs sur le sujet

Ce qui réunit les habitants d'une collectivité territoriale, c'est une géographie. Pour les membres d'une association sportive, d'une fédération, c'est une passion.

arguments, la parité ne serait pas un objectif, elle serait simplement subie. Pour notre part, nous voulons en faire un objectif. L'amendement du Gouvernement, même s'il va dans le bon sens,

parole est à Mme la ministre déléguée. Il y a presque dix ans, la loi pour l'égalité réelle entre les femmes et les hommes instaurait, pour la première fois, un objectif de représentation équilibrée des femmes et des hommes dans les instances dirigeantes des fédérations sportives.

a financé des plans de féminisation des fédérations. Nous avons financé aussi le programme « dirigeantes » du CNOSF, et plusieurs fédérations se sont investies pour mobiliser leur territoire et instaurer des mécanismes de parité au sein de leurs instances sportives. Depuis 2017, le Président de la République a fait de l'égalité femmes-hommes la grande cause de son quinquennat.

exceptionnelle, à la tête des plus grandes instances sportives, sont d'accord pour aller dans ce sens. Elles m'ont confirmé leur soutien pour le projet d'une parité totale dans les instances fédérales d'ici à 2024.

C'est pourquoi nous proposons qu'au niveau régional, cette date soit reportée à 2028, non parce que nous serions moins ambitieux, mais parce que les organes régionaux sont élus avant les organes nationaux. Cela donnerait la possibilité,

cohérents. On ne peut pas vouloir la promotion du sport féminin et, en même temps, se détourner de la question de l'égalité hommes-femmes dans la gouvernance du sport. Il y a

de porter à 50 % la représentation minimale de chacun des deux sexes dans les instances dirigeantes des fédérations et d'étendre cette représentation minimale aux instances dirigeantes des organes déconcentrés régionaux des fédérations qui délivrent plus de 25 % des licences à l'un des deux sexes, le tout avec une période transitoire de dix-huit

Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement. Le scrutin est ouvert.

de la commission ? Une telle disposition pourrait avoir pour effet de renforcer la tendance actuelle à faire évoluer les fédérations et les ligues vers un statut d'organisateurs de spectacles, en contradiction avec

que ces associations peuvent affilier. Il s'agit de personnes physiques- les supporters peuvent évidemment en faire partie -, de structures commerciales ayant ou non pour objet la pratique sportive ou son développement, et des clubs professionnels. Les associations ou les groupements de supporters peuvent donc déjà se voir accorder la qualité de membres des fédérations. Beaucoup de fédérations ont créé des clubs de supporters, notamment autour de leurs équipes de France. Je fais confiance aux fédérations ou aux ligues professionnelles pour s'emparer de l'enjeu de la fidélisation des supporters,

le critère de la capacité à participer à la mise en oeuvre de la politique du sport apparaît insuffisamment précis et opérationnel. Cependant, l'amendement vise- vous l'avez rappelé -à répondre au problème que peut rencontrer le mouvement sportif lorsque certaines fédérations se retrouvent en déshérence et doivent être restructurées ou rapprochées.

aux personnes en situation de handicap. La commission du Sénat a supprimé cet article, tout en saluant son objectif, précisant dans son rapport que nombre de fédérations délégataires ne pourraient pas proposer de tels programmes, faute d'équipements ou d'expertise adaptée, et que cette généralisation ne présentait aucune garantie de qualité dans l'accueil et la prise en charge. Nous sommes d'accord sur le constat, mais pas sur la conclusion : si le principe peine à s'appliquer, c'est justement parce que nous manquons de moyens pour le faire appliquer. Dans ce cas, investissons ! Donnons des moyens

notamment au regard du déséquilibre important entre le nombre d'associations et celui des structures professionnelles. Il nous semble que l'on pourrait généraliser ce modèle, en posant un principe simple : les associations qui représentent l'essentiel des acteurs du quotidien, et qui sont au centre de la politique sportive, doivent être majoritaires au sein de l'organe dirigeant de la discipline sportive. C'est d'autant plus légitime à nos yeux qu'il s'agit en fait du seul lieu de gouvernance dont elles disposent, à la différence des clubs professionnels, qui sont eux réunis dans les ligues professionnelles. En l'état, la proposition de loi que nous examinons franchit déjà un premier pas intéressant, puisqu'elle prévoit la parité entre ces deux structures dans les instances. Mais il nous semble qu'on pourrait aller plus loin en accordant une petite majorité aux associations.

réserver 50 % des voix aux représentants des associations et aux membres de la fédération. Nous proposons donc, de façon raisonnable et proportionnée, de limiter les postes réservés au sein des instances dirigeantes des fédérations, en prévoyant qu'ils ne devront pas excéder 25 % des sièges.

qu'une association des athlètes de haut niveau. C'est un premier pas qu'il faut saluer, mais, notamment pour une question de parallélisme des formes, il apparaît indispensable que cette facilité soit aussi accordée aux arbitres et juges sportifs de haut niveau. Ces derniers font vivre le sport et les valeurs sur le terrain et dans les compétitions ; il est donc tout à fait légitime qu'ils siègent dans les conseils directeurs. De nombreuses fédérations n'ont d'ailleurs pas attendu cette loi pour les y associer.

établissent des listes électorales mixtes comprenant déjà des arbitres et des juges en leur sein. Il convient de conserver une certaine souplesse dans les modes de désignation afin de ne pas faire peser sur les fédérations des obligations trop importantes, lesquelles bouleverseraient inutilement une vie démocratique interne qui fonctionne.

Mme Béatrice Gosselin. Cet article précise les modalités de participation des athlètes de haut niveau à la vie démocratique des fédérations. Cette évolution est parfaitement justifiée, mais il convient de préciser que les arbitres et les juges sont eux aussi essentiels à la pratique sportive. Sans eux, pas de compétition ni d'éducation à la règle sportive. Le dispositif proposé par cet amendement permet un parallélisme des formes avec les dispositions applicables aux athlètes afin que les voix des 246 000 arbitres et juges sportifs de notre pays, gardiens des règles du jeu, puissent s'exprimer, l'arbitrage sportif est frappé par une crise des vocations sans précédent, cet amendement est à la fois gage d'écoute et de reconnaissance pour les juges et les arbitres sportifs, qui ne doivent pas être les oubliés de la vie sportive. L'amendement n° 27, présenté

est une réelle avancée pour reconnaître leur rôle dans la politique sportive du pays. Mais c'est oublier un peu vite les arbitres et juges, pourtant indispensables à la pratique sportive. On ne peut décemment concevoir que ces derniers soient totalement exclus des instances dirigeantes des fédérations,

ou en aval. Madame la ministre, mes chers collègues, il est minuit. En accord avec la commission et le Gouvernement, je vous propose de prolonger notre séance jusqu'à une heure du matin pour poursuivre l'examen de ce texte. Il n'y a pas d'observation ? ... Il en est ainsi décidé.

à rendre spécifique le choix de ces athlètes pour les sports professionnels où il existe un dialogue de branches entre le syndicat des joueurs et des joueuses

Cet amendement vise à fixer une obligation de moyens aux fédérations sportives pour informer leurs licenciés sur l'existence d'une assurance protection juridique et psychologique en matière de violences sexuelles.

de l'être à l'avenir, en faisant en sorte que les fédérations, au même titre qu'elles invitent leurs adhérents à souscrire une assurance individuelle accident,

l'article 6 issue de l'Assemblée nationale et l'ajout de notre rapporteur. Cet article, relatif au rôle du CNOSF en matière de déontologie sportive, prévoyait à l'issue des débats à l'Assemblée nationale à l'Assemblée nationale la réalisation par celui-ci d'un rapport concernant l'inclusion de tous les publics ainsi que la lutte contre les discriminations et les violences physiques, sexuelles et sexistes. Il prévoyait aussi d'inclure dans la charte du CNOSF la démarche des objectifs de développement durable de l'ONU. En commission, notre rapporteur a fait voter une réécriture qui revient peu ou prou à la formulation actuelle de l'article L. 141-3 du code du sport. L'ajout du terme

et écologique de l'Assemblée nationale et l'apport de notre rapporteur. L'amendement

Au cours de ces dernières années, les violences sexuelles et sexistes ont été particulièrement mises en lumière dans plusieurs disciplines. On ne peut toutefois ignorer l'important travail entrepris par le Gouvernement pour lutter contre toutes les formes de violences et de discriminations. L'article 6 permettra d'accompagner un peu plus cette politique s'il est assorti d'une demande imposant au CNOSF de produire un rapport public valorisant notamment son action pour l'inclusion de tous les publics, la lutte contre les discriminations et contre les violences physiques, verbales et sexuelles.

particulièrement attentifs aux problématiques d'éthique. L'un de nos anciens membres, Yvon Collin, fut d'ailleurs à l'origine de la loi de 2012 visant à renforcer l'éthique du sport et les droits des sportifs. Quel est l'avis de

n° 79 rectifié. Cet amendement vise à limiter à trois le nombre de mandats des présidents de fédérations sportives agréées, comme le prévoyait initialement le texte transmis par l'Assemblée nationale. Pourquoi avoir supprimé une telle mesure, alors que les usages en cours dans le sport ou ailleurs tendent à converger vers le principe d'une limitation des mandats ?

nous proposons, en cohérence avec nos convictions et dans le respect de l'aspiration démocratique des pratiquants, de rétablir la limitation dans le temps des mandats de président de fédération sportive. L'amendement n° 104

Le dispositif est en train de se mettre en place. De nouvelles présidentes arrivent à la tête de fédérations. Peut-être cela ne va-t-il pas assez vite, mais le processus est engagé

du 1 mars 2017 visant à préserver l'éthique du sport, à renforcer la régulation et la transparence du sport professionnel et à améliorer la compétitivité des clubs. Quel est l'avis du Gouvernement ? Monsieur le

le tissu associatif a considérablement souffert ces dernières années de la réduction drastique du nombre d'emplois aidés. Au travers de la présence d'un tel

à la situation difficile qu'elles vivent. Avoir un référent sur ce thème ne nous paraît pas utile, dans la mesure où nous discutons directement avec les acteurs associatifs. Ainsi, quand des fédérations désirent se saisir du sujet, nous les incitons à passer des partenariats

Sur un sujet aussi grave que celui des viols sur mineurs, il me semble important d'obliger les fédérations à faire preuve de volontarisme. Ainsi, le présent amendement tend à rendre obligatoire la nomination d'un référent aux violences sexuelles au sein de chaque fédération sportive. Quel est l'avis de

La prévention de toutes les formes de discrimination est l'un des combats sociétaux de notre jeunesse, l'une des luttes des XX et XXI siècles. Le sport est un langage universel qui unit les peuples à travers le jeu, quels que soient les acteurs et les actrices, leur niveau technique, l'équipement et les moyens disponibles. Il subsiste malheureusement, dans les enceintes sportives, encore des comportements violents, des haines qui peuvent s'exprimer, des atteintes à l'honneur ou à la dignité humaine. Ces comportements doivent être combattus par tous les moyens juridiques disponibles, notamment les actions judiciaires que peuvent engager les associations de défense des droits humains. Cet amendement vise à compléter l'article L. 332-17 du code du sport, afin de permettre à toutes les associations qui luttent contre les discriminations portant sur l'identité des personnes d'exercer les droits reconnus Il s'agit de permettre ainsi à toute personne victime d'une discrimination en raison de son sexe, de son orientation sexuelle ou de son handicap de bénéficier, au cours de la procédure, de l'accompagnement d'une association spécialisée, comme cela est déjà le cas en matière de discrimination à caractère raciste, xénophobe et antisémite.

Cet amendement tend à prévoir, au titre de peine complémentaire pour les personnes jugées coupables d'incitation à la haine ou à la violence discriminatoire lors d'une manifestation sportive, la possibilité d'accomplir un stage de sensibilisation à la lutte contre les discriminations.

aucune indication n'est fournie sur sa durée, son organisation, son coût et son contenu. La mise en oeuvre de cette disposition ne me paraît donc pas très assurée. L'avis est défavorable.

à caractère régional ou d'y participer. L'article 8 , tel qu'il était rédigé, répondait à une ancienne et forte demande du monde sportif ultramarin. L'enjeu ici n'est pas de créer les conditions d'un fédéralisme institutionnel. Toute l'ambition de cette disposition est de donner aux athlètes ultramarins, souvent jeunes, les moyens de s'entraîner et de concourir dans leurs bassins régionaux respectifs. Nous proposons donc de revenir à la rédaction initiale de cet article.

monsieur le rapporteur, rédaction proposée par l'Assemblée nationale en ajoutant seulement une référence à la nécessité d'un accord préalable de la fédération nationale. Pour autant, à nos yeux, tous les risques ne sont pas levés. La rédaction de l'amendement évoque toujours l'affiliation des ligues et comités sportifs à une fédération régionale, ce qui ouvre la porte à une forme d'indépendance de ces structures à l'égard à l'égard de la fédération nationale, puisque la notion d'affiliation crée un lien de subordination. Par ailleurs, on comprend mal comment une équipe pourrait concourir, à la fois, au nom de la France et au nom de la collectivité à laquelle elle appartient. Quelles seraient, par ailleurs, les sanctions en cas de manquement à

qui permettent aux licenciés optant pour cette solution de pratiquer plusieurs activités à un tarif plus avantageux que celui découlant de la prise de deux, trois ou quatre licences. Ce dispositif permettrait de favoriser le développement de la pratique sportive pour le plus grand nombre et d'inciter les personnes à essayer la pratique de sports différents avant, éventuellement, de s'orienter vers un choix définitif.

Les droits de diffusion audiovisuelle sont la première source de financement du sport professionnel. En France, le marché des droits de diffusion est aujourd'hui estimé à 1,8 milliard d'euros. Une partie de ces recettes revient au sport amateur en application du principe de solidarité, de solidarité, laquelle s'exerce par l'intermédiaire de la taxe Buffet. L'État prélève ainsi 5 % du produit des droits de diffusion pour les affecter à l'Agence nationale du sport et au budget de l'État. Cette solidarité s'exerce également au sein des fédérations, qui sont tenues de reverser une partie du produit des droits au développement de leur secteur amateur. Par exemple, la Ligue de football professionnel reverse chaque année 2,5 % du produit des droits à la Fédération française de foot. Le sport amateur ayant durement souffert de la crise sanitaire, avec la chute du nombre de licenciés et la fragilisation du bénévolat, un relèvement de la taxe Buffet, qui, en outre, peut pâtir d'un rendement aléatoire, permettrait de mieux sécuriser le soutien, plus que nécessaire, au sport amateur.